En renvoyant la définition du minimum de pension à l'hypothétique future réforme systémique des retraites, le Gouvernement compromet la mise en oeuvre immédiate de la mesure principale de ce texte : madame la ministre ! Cette méthode

souligné, les conséquences de ces pratiques sont désastreuses pour notre économie et nos politiques publiques ; le consentement à l'impôt, qui fonde notre pacte républicain, s'en trouve gravement affecté.

Ces travaux, dont l'initiative revient à quelques États, dont la France, ont été conduits sur demande du G20 et dans le cadre de l'OCDE au titre du chantier, des mesures opérationnelles